Il vous est demandé de laisser un siège vide entre deux sièges occupés. J'invite chacune et chacun à veiller au respect des distances de sécurité. Je rappelle également que les sorties de la salle des séances devront exclusivement s'effectuer par les portes situées au pourtour de l'hémicycle. J'informe le Sénat que les commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure, du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, ne sont pas parvenues à l'adoption de textes communs. En conséquence, les lectures des conclusions des commissions mixtes paritaires sur ces textes, préalablement inscrites à l'ordre du jour du mardi 27 octobre et du mercredi 4 novembre, sont retirées de l'ordre du jour. Il appartiendra au Gouvernement de demander l'inscription de l'examen de ces textes en nouvelle lecture à l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat. M. Bernard Buis, élu juge suppléant à la Cour de justice de la République le 21 octobre dernier, va être appelé à prêter, devant le Sénat, le serment prévu par l'article 2 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République. Je vais donner lecture de la formule du serment. je vous prie de bien vouloir vous lever et de répondre, en levant la main droite, par les mots : « Je le jure jure ». Voici la formule du serment : « Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Acte est donné par le Sénat du serment qui vient d'être prêté devant lui.

Dans la discussion générale, la parole est à M. Laurent Lafon, auteur de la proposition de loi. Monsieur

Tout l'objet de cette proposition de loi est de renforcer l'information des citoyens. Il est donc essentiel que le diagnostic de cybersécurité aboutisse à un dispositif coloriel, présenté aux Français lors de chaque connexion au service. Le Cyberscore ne doit surtout pas être relégué dans les abîmes des conditions générales d'utilisation, ce qui reviendrait à vider la proposition de loi de sa substance.

économiques, éducatives et médicales seront bouleversantes. La certification que prévoit ce texte répond aux attentes formulées par les acteurs économiques français du numérique. Rassemblés autour de la plateforme Mailo, ils ont signé en juillet dernier une tribune appelant à la création d'un label

à faire émerger plus rapidement des services alternatifs aux géants du numérique américains et chinois. Chaque utilisateur qui se connecte à ces plateformes leur livre une matière première dont il ne perçoit pas nécessairement la valeur économique. L'émergence d'une filière numérique européenne est donc indispensable.

Elle s'intéresse tout particulièrement à la sécurité des données, personnelles ou non, c'est-à-dire à l'ensemble des traces que nous laissons sur internet.

La crise du covid a certes amplifié les fractures numériques, sociales, territoriales ou financières qui isolent près de 13 millions de nos concitoyens, mais elle a aussi fait exploser certains usages, dont les commandes en ligne et les visioconférences, à des fins tant professionnelles que personnelles.

Selon un sondage, 90 % des Français considèrent que les données personnelles sont précieuses et qu'elles devraient être davantage protégées. Ils sont aussi conscients qu'elles sont convoitées par les géants du Net. Pour autant, cette prise de conscience n'entraîne pas systématiquement de changement dans les pratiques. Or, en recourant à des plateformes plus ou moins sécurisées, les consommateurs s'exposent à des risques, enregistrement vidéo à l'insu des participants, utilisation de la reconnaissance vocale, attribution de propos qu'on pense oubliés, espionnage, ... Les Les pouvoirs publics sont eux aussi la cible grandissante d'attaques, en particulier les collectivités territoriales et le secteur de la santé. Par conséquent, au-delà de la menace permanente des cyberattaques dont il faut se protéger,

La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui comporte deux articles, dont le premier concerne l'information des consommateurs, et le second celle des acheteurs publics. L'article 1 prévoit de créer un dispositif nommé Cyberscore, par référence au Nutriscore.

Cette disposition comble un vide dans les textes qui encadrent actuellement la cybersécurité des solutions numériques. Elle devrait être compatible, voire complémentaire, de la stratégie de cybersécurité en cours d'adoption au niveau européen. Nous avons adapté le dispositif aux services les plus utilisés, selon des seuils à déterminer par le pouvoir réglementaire. Il ne pèsera donc pas sur l'innovation et ne sera pas non plus un frein au déploiement de jeunes pousses du numérique. Il se veut souple et réactif aux évolutions technologiques, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de définir des indicateurs de mesure

Les indicateurs fournis pourraient même aller jusqu'à intégrer des paramètres de lutte contre la haine en ligne. Avec l'accord de Laurent Lafon, nous proposerons quelques amendements

Cependant, force est de constater que les choses évoluent et que ces risques sont de mieux en mieux appréhendés. Les scandales de fuites de données chez des géants du numérique, tels que Facebook, Uber ou Yahoo, font ainsi régulièrement la une de l'actualité.

Apporter une réponse systémique- je le dis -, c'est le sens des travaux que mène la France, mais aussi de ceux qui sont en cours au niveau européen. Ils visent à faire émerger des lignes fortes, solides et transnationales, de nature à assurer au mieux notre souveraineté numérique. Comme pour le RGPD, l'Europe doit se montrer à la hauteur des enjeux et définir ses propres standards,

Les ajouts proposés par le Gouvernement concernent également le champ d'application du dispositif, afin de le restreindre, dans un premier temps, aux plateformes de taille mondiale, soit les acteurs auprès desquels il est le plus important d'intervenir. Enfin, ces changements concernent l'inscription dans le code de la commande publique, qui ne me semble pas être la voie la plus efficace pour agir : j'y reviendrai.

Je vous remercie

pour objectif de mieux informer les consommateurs sur le niveau de sécurité des services qu'ils utilisent. La commission des affaires économiques a introduit un mécanisme de score qui a l'avantage d'apporter plus de clarté, il me semble d'ailleurs que cela est assez symptomatique : le sujet n'est pas lisible. Hormis certains spécialistes, très peu d'entre nous connaissent le fonctionnement des outils numériques. Nous savons les utiliser- les concepteurs veillent d'ailleurs à produire des logiciels très ergonomiques -, mais nous ignorons les principes qui régissent ce monde particulier, encore naissant à bien des égards. L'information du public sur les risques est une avancée qu'il nous faut soutenir. Elle implique toutefois un travail important, parce qu'il sera nécessaire d'établir, mais aussi de mettre à jour, ces diagnostics cela exigera des efforts prolongés. Pour améliorer l'information des consommateurs, nous devrons également développer l'enseignement du numérique, à l'école et hors de l'école.

Les responsables de la sécurité des systèmes d'information sont encore trop nombreux à plaisanter en affirmant que la plupart des failles se situent « entre la chaise et le clavier » ; sans une bonne connaissance de l'outil, il est difficile de se prémunir contre les

... Sans nous condamner à un retour à l'âge de pierre, les spécialistes de la cybersécurité font de la résilience l'une des composantes essentielles de la défense. En effet, personne n'étant immunisé contre une cyberattaque, il s'agit de savoir se relever lorsque l'agression a réussi. Tout comme l'évaluation du risque et les moyens d'y faire face, la résilience implique de développer une culture numérique. L'usager doit être averti des pièges à éviter et être conscient des failles ; cela n'est possible qu'avec une bonne connaissance du milieu. Le cyberespace est un espace à part entière, où les enjeux sont multiples souveraineté, extraterritorialité, sécurité des personnes dans la gestion de leurs données et protection de la vie privée. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus dépendants de services numériques souvent étrangers. Il est donc urgent de maîtriser pleinement cet outil, avant qu'il ne soit trop tard.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons cet après-midi la proposition de loi pour la mise en place d'une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public. cette proposition de loi, on cherche à répondre aux craintes légitimes, exprimées pendant le confinement, sur le traitement de nos données personnelles collectées les outils et autres plateformes de visioconférence facilitant le télétravail. Tout d'abord, je me réjouis que la problématique de l'exploitation des données personnelles soit à l'ordre du jour du Sénat. Voilà un sujet majeur, qui touche aux questions de transparence et d'information du consommateur internaute sur la sécurisation de ses données et aux questions de souveraineté numérique, tant en France qu'à l'échelon européen. Si l'évolution des technologies permet aujourd'hui une expansion bienvenue du télétravail, nous devons sensibiliser nos concitoyens à ces enjeux de cybersécurité et rappeler que la pratique du numérique conduit à s'exposer à un certain nombre de risques. Ainsi, les internautes, mais aussi les entreprises, sont particulièrement sujettes aux risques et doivent encore, pour une large majorité d'entre elles, s'approprier certains réflexes. À l'heure où le numérique est partout et où le Gouvernement pousse au déploiement, sans débat et sans concertation, de la 5G, rappelons que la vigilance et la tempérance dans les pratiques et les usages du web sont primordiales pour ne pas exposer nos concitoyens ni aggraver notre bilan carbone. Si de nombreux textes, à commencer par le RGPD, cette proposition de loi représente un pas supplémentaire vers plus de transparence et de droits pour les internautes, ce qui va évidemment dans le bon sens. Nous soutenons donc la principale mesure de ce texte la mise en place d'un Cyberscore, un diagnostic de cybersécurité lisible, clair et compréhensible par tous. Je m'interroge néanmoins sur la portée de l'amendement de Mme la rapporteure adopté en commission étend le champ d'application du dispositif à tous les services numériques, notamment aux logiciels de visioconférence, elle limite le champ d'application aux services numériques les plus utilisés, selon des seuils à définir. La commission a justifié cet aménagement en indiquant que cela « évitera d'imposer de trop fortes contraintes à de petites structures », mais nous pensons au contraire que les petites entreprises du numérique ont tout à gagner à faire valoir la fiabilité de leur plateforme et à faire respecter une gestion responsable C'est justement une belle occasion pour elles de se démarquer des géants du numérique, qui ne sont pas toujours exemplaires en la matière. En outre, nous pensons également que c'est un pli à prendre pour toutes les nouvelles entreprises qui se lanceront dans ce secteur. Nous souhaitons par ailleurs alerter la Haute Assemblée de l'amendement qu'a déposé le Gouvernement sur l'article 1. Cet amendement tend à atténuer largement la portée de cet article, notamment en retirant l'obligation d'une évaluation des plateformes par une autorité administrative indépendante

Nous devons aller plus loin encore, notamment dans le cadre d'une évolution du RGPD. En effet, c'est bien évidemment à l'échelon européen que la démarche globale de certification de cybersécurité doit s'engager et avancer. Des évolutions récentes ont été actées, avec le ; la France doit maintenant rapidement s'approprier ce chantier de la certification. Dans un monde numérique dominé aujourd'hui par les grands acteurs américains et chinois, notre souveraineté nationale dépend de l'Europe, tout comme l'Europe a besoin de la France pour se développer dans ces domaines. Nous disposons de tous les outils pour y parvenir : la technologie, le savoir-faire, une main-d'oeuvre hautement qualifiée. Il faut être à l'avant-garde de ces enjeux d'avenir, mais il faut aussi garder une lucidité pleine et entière pour analyser les avantages et les inconvénients de la numérisation de la société. La parole

si le confinement a eu une vertu, c'est celle de nous montrer à quel point les Français pouvaient, malgré leurs privations de liberté, faire preuve d'imagination, de créativité, de réactivité et de résilience pour briser les barrières physiques que nous imposaient les règles sanitaires. Télétravail, télémédecine, visioconférence, sport en ligne, représentations artistiques : c'est en grande partie grâce au numérique que ces solutions de remplacement salvatrices ont pu s'exprimer. L'écosystème français a donc dû s'adapter à ces nouvelles règles, grâce au numérique, qui connaît en France une certaine maturité : notre pays compte en effet 53 millions d'internautes mensuels, ce qui représente 92 % de foyers connectés dans l'Hexagone. Bloqués à leur domicile pendant deux mois, les Français n'auront jamais autant utilisé internet que pendant la période de confinement. Par exemple, en avril 2020, les trois quarts des Français, soit 46 millions de personnes, se sont connectés tous les jours.

jour. Or la sécurité requise dans l'espace public vaut aussi pour l'espace numérique. L'ensemble de notre quotidien, personnel et professionnel, repose un peu plus chaque jour sur des outils et plateformes numériques susceptibles d'utiliser nos données personnelles en vue d'actes malveillants. malveillants. Le nombre d'attaques en ligne ne cesse d'augmenter. Dans ce contexte, le travail de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui assure un service de veille, de détection, d'alerte et de réaction aux attaques informatiques, notamment sur les réseaux de l'État, est crucial. Néanmoins, au regard des menaces grandissantes, il paraît nécessaire que cette agence soit renforcée par de nouveaux moyens humains et structurels.

en 2019, l'Anssi n'avait compté que 54 cas. C'est donc déjà deux fois plus, alors que l'année n'est pas encore finie ... Face à cette insécurité qui progresse de façon exponentielle, il ne fait pas de doute que nous accueillons cette proposition loi avec bienveillance. article 1 propose que les consommateurs soient mieux informés sur la sécurisation des données lorsqu'ils utilisent solutions numériques, l'objectif étant de mettre place, à terme, une sorte de Nutriscore de la cybersécurité. Nous ne pouvons que souscrire à cette proposition. Il faudrait toutefois que les modalités du diagnostic soient précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés du numérique et de la consommation, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL ; tel est l'objet d'un amendement du Gouvernement. Cela montre également qu'un travail coconstruction entre la rapporteure et le Gouvernement a pu être mené pour aboutir à un texte aussi efficace que techniquement réalisable. la rapporteure souhaite intégrer, parmi les fournisseurs de service en ligne, les acteurs de services de visioconférence en ligne, particulièrement sollicités dans cette situation sanitaire particulière, notamment pour le télétravail. Il est vrai que nous n'avons que peu d'informations sur le stockage des données de ces plateformes, qui s'accommodent assez facilement du règlement européen sur la gestion des données, auxquelles elles doivent se soumettre. Il nous paraît donc assez cohérent de souscrire, au premier abord, à l'idée d'un tel sous-amendement.

ce projet de Cyberscore nous paraît-il particulièrement bienvenu pour répondre aux nombreuses interrogations des internautes. Nous voterons donc cette proposition de loi. La parole est à M. Jean-Claude Requier. Monsieur

ce texte, issu de la commission des affaires économiques, s'inscrit dans la série de travaux réalisés par le Sénat, depuis un certain temps, dans le domaine du numérique et des technologies de l'information. Ainsi, rappelons la proposition de loi adoptée en début d'année visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace, la question du statut des travailleurs de plateforme,

enjeu de longue date, est une question encore plus centrale depuis les mesures de lutte contre la pandémie de covid-19 et le recours massif au travail à distance, au moyen d'outils numériques. le confinement a accéléré l'utilisation de ces outils, à des fins tant professionnelles que privées. Dans ce contexte, le recours, parfois dans l'urgence, à des applications de téléconférence n'est pas allé sans augmenter les risques de piratage, d'enregistrement indu ou de détournement de données personnelles. Je fais également remarquer que les collectivités territoriales, ne bénéficiant souvent pas des mêmes ressources que l'État, sont plus vulnérables à la cybercriminalité. l'initiative du groupe UC et de notre collègue Laurent Lafon procède d'une intention légitime : renforcer la sécurité des plateformes numériques, en particulier des outils de téléconférence et de commande en ligne, en instaurant une obligation de certification. Concrètement, les services de communication en ligne devront communiquer les informations relatives à la sécurité des données hébergées par eux ou par un autre prestataire. Cette démarche devra néanmoins s'articuler avec, d'une part, les travaux en cours à l'échelon européen, et, d'autre part, les aspects relevant du domaine réglementaire. Si la pertinence du sujet ne fait pas de doute, le véritable enjeu se trouve dans sa technicité et dans l'applicabilité de nouvelles dispositions : champ d'application de la certification, niveau adéquat de norme, effectivité face à des acteurs de niveau mondial. du RDSE souscrit en principe à cette initiative. Je me permets simplement d'exprimer une réserve ou, du moins, une interrogation sur les éventuelles conséquences financières de cette nouvelle obligation. La certification sera-t-elle payante ? Les start-up et autres petites entreprises n'ont pas forcément les moyens de remplir ce type d'obligation, ce qui risque de créer une concurrence déloyale avec les plus grands acteurs. La rapporteure a assuré que la modification adoptée en commission la semaine dernière les protégera de ce risque, mais elle renvoie à un décret pour la définition des seuils d'utilisation. Or on sait que les décrets prennent parfois du temps à être adoptés Combien de temps faudra-t-il attendre pour obtenir le précieux sésame ? En conclusion, le groupe du RDSE salue cette initiative dans un domaine pleinement d'actualité, où les risques d'abus sont généralement sous-estimés.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, de nombreux enjeux éthiques, démocratiques et économiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont directement liés à l'essor des nouvelles technologies et à la généralisation de l'utilisation d'outils informatiques et numériques. À l'ère de l'omniprésence de l'informatique et des objets connectés, la question de la sécurité des systèmes est donc centrale. Aussi, en matière de cybersécurité, deux axes nous semblent essentiels. La première problématique est celle de la cybercriminalité et des piratages. En effet, 80 % des entreprises disent avoir été touchées par au moins une cyberattaque en 2018. Le pire est que l'on observe à la fois une professionnalisation des cyberattaquants et une multiplication des cyberdélinquants. À cet égard, l'explosion du télétravail, en cette période de crise sanitaire, a mis en lumière la fragilité des particuliers des cyberdélinquants. À cet égard, l'explosion du télétravail, en cette période de crise sanitaire, a mis en lumière la fragilité des particuliers et de nombreuses entreprises. Plusieurs questions se posent : pourquoi mes données personnelles doivent-elles être protégées ? Que se passerait-il si nos objets numériques partageaient librement nos données avec un tiers ? Que pourrait en faire ce dernier ? Et les mêmes interrogations se posent pour une entreprise, pour un service public ou pour un État. par les usagers, de connaissances sur la cybersécurité et une meilleure information sont une nécessité, il n'en demeure pas moins que c'est d'un véritable effort de formation que nous avons besoin, d'autant que la France fait face à une pénurie de cyberspécialistes. De nombreux objets connectés d'un usage quotidien ne sont souvent que très faiblement sécurisés, alors même qu'ils pénètrent dans les foyers et sont susceptibles de donner accès à toutes sortes d'informations sensibles. exemples récents : la découverte, dans un robot-cuiseur, d'un micro, dont aucune mention n'était faite dans la notice, ou encore les Vtech Leaks, en 2015, avec le piratage de plus de 6 millions de comptes de tablettes pour enfants, qui était, fort heureusement, le fait d'un militant souhaitant démontrer la non-fiabilité de ces appareils. Ajoutons à cela l'étude de chercheurs de l'université de l'Iowa, qui ont trouvé une douzaine de failles de sécurité que la 5G pourrait aggraver, sans qu'il soit nécessaire, pour les pirates, de disposer d'un équipement de pointe. À toutes ces questions sociétales, commerciales et économiques, on pourrait ajouter des problématiques de défense nationale, alors même que le cyber fait partie des nouveaux champs de bataille de la guerre hybride. La deuxième problématique à laquelle nous devons faire face est l'extraterritorialité des lois états-uniennes, qui permettent au gouvernement des États-Unis de demander, en justice, l'accès à toute donnée personnelle détenue par une entreprise américaine, où qu'elle soit implantée dans le monde. monde. Rappelons-le, aux États-Unis, le secret professionnel n'existe pas face à la raison d'État. Il est donc impératif, en cas de marché public, de prendre en compte ces risques. D'ailleurs, le 16 juillet dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a cassé l'accord sur les données personnelles passé entre les États-Unis et la Commission européenne, considérant que ce traité ne protégeait pas suffisamment les citoyens européens. Le risque est que, avec le, les données publiques sensibles tombent sous le coup de la législation états-unienne. C'est notamment le cas pour ce qui concerne les données de santé, qui devaient être hébergées dans les de Microsoft, aux Pays-Bas. Or Microsoft étant une société américaine, elle est soumise au des États-Unis. Qui plus est,

pour l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, le développement des technologies de l'information et des communications est de plus en plus difficile à encadrer. Permettre le développement du numérique, tout en garantissant la sécurité, la protection des données et la confiance des consommateurs, est un défi difficile à relever. Ce débat est l'occasion de le rappeler, le déploiement d'un parcours d'identification numérique, au travers duquel chaque citoyen pourra prouver son identité en ligne, dépend aussi de la capacité de chaque usager à s'approprier de tels systèmes, aussi intelligents soient-ils. Cette capacité dépend directement du degré de confiance qu'auront ces usagers à l'égard des plateformes numériques. L'actualité montre à quel point nous sommes devenus vulnérables face à un nouveau modèle, qui s'impose implacablement. Il faut apprendre à vivre dans ce monde où chaque instant de notre vie devient perméable à toutes sortes d'intrusions, en raison du développement des objets connectés. Même au siècle de l'intelligence artificielle, personne ne peut contester le fait que le risque zéro n'existe pas. Les failles existeront toujours, et les victimes doivent être prises en charge. C'est une question tant juridique,

Aussi, la question des données personnelles des citoyens doit être au coeur de nos préoccupations. La protection de ces derniers doit être renforcée, notamment dans le cadre d'une évolution du RGPD, Il faut améliorer le dispositif de consentement des utilisateurs et mieux alerter ceux-ci quant aux risques liés à l'exploitation de leurs données. Cette réflexion doit être menée rapidement, dans le cadre d'une approche qui englobe la question de la neutralité des réseaux et des terminaux, la portabilité des données et l'interopérabilité des plateformes. Le Sénat a beaucoup travaillé ces derniers mois sur ces sujets, qu'il s'agisse du rapport sur la souveraineté numérique proposition de loi visant à renforcer le droit des consommateurs dans le cyberespace, adoptée à l'unanimité dans cet hémicycle, mais l'appropriation de cette question par le grand public doit être renforcée.

lui-même. À l'article 1, le Cyberscore, issu des travaux en commission et équivalent à un Nutriscore de la cybersécurité des solutions numériques, aura le mérite d'apporter aux utilisateurs un repère simple, pour

devrait figurer lors de chaque connexion au service, à l'image du diagnostic de performance énergétique. La version proposée par le Gouvernement nous convient, d'autant qu'elle inclut la consultation de la CNIL sur les indicateurs qui seront pris en compte par le diagnostic de cybersécurité. Elle satisfait donc l'amendement que nous avions déposé initialement. Il est également indispensable que l'ensemble des opérateurs de service de communication en ligne soit concerné, et non pas seulement les plateformes numériques. Nous voterons donc pour le sous-amendement de la rapporteure, afin d'inclure, dans le champ de la proposition de loi, les éditeurs d'application de visioconférence, par exemple. Dans un monde de réseaux, où l'information circule de plus en plus rapidement, il est indispensable de garantir aux acteurs publics la sécurité de leurs données stratégiques. Il s'agit donc de protéger leur développement et leur transformation numérique. Les collectivités territoriales, par exemple, traitent un volume croissant de données personnelles, afin d'assurer le fonctionnement des services publics dont elles ont la charge. La divulgation de ces données- fiscales, sociales ou autres -, leur altération, leur suppression ou leur vol constituent des atteintes dommageables en soi, elles ont également de graves répercussions sur le déroulement du processus de modernisation de l'administration et des services des collectivités visées.

La présence d'un écosystème dédié sur un territoire, composé de et complété par des PME et des start-up, ainsi que par la présence d'une offre de formation, sont autant d'atouts pour favoriser le développement de la filière sur les territoires et l'accueil de nouvelles entreprises.

Je rejoins les différents orateurs pour souligner la nécessité de ne pas laisser les consommateurs démunis face aux solutions numériques qu'ils utilisent. La solution d'un Cyberscore, proposée ici, me paraît, ainsi qu'à l'ensemble de la commission des affaires économiques, particulièrement pertinente.

vous connaissez mon attachement à la défense du consommateur dans le cyberespace. Aussi, je ne manque pas l'occasion de rappeler que cette protection du consommateur passe également, à notre sens, par un encadrement plus structurel des pratiques des géants du numérique. Ces pratiques tendent à enfermer le consommateur dans un web en silo, à rebours du web eldorado des libertés et des opportunités. Ce matin, en commission mixte paritaire, nous ne sommes pas parvenus à un accord sur ce sujet : alors qu'une majorité se dessinait clairement, le Gouvernement a donné l'ordre à sa majorité de renoncer à toute ouverture

Nous avons donc une vision différente de la défense du consommateur. J'ajoute que nous avions proposé de reporter à 2023 la mise en application des dispositifs adoptés deux fois à l'unanimité par le Sénat, afin de vous permettre de mener les négociations européennes et d'avoir des solutions nationales

alors qu'il reconnaît la nécessité d'une législation européenne. Le Gouvernement semble donner ici un gage de sa volonté d'avancer sur ce point relatif à l'information du consommateur, même si tout dépend encore de l'inscription du texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Nous verrons donc ... Cette proposition de loi me donne l'occasion d'évoquer la question de la sécurisation des données de nos entreprises, en particulier de leurs données stratégiques. la confidentialité de ces données peut être fragilisée par des lois de portée extraterritoriale. Au travers d'initiatives comme Gaïa-X, les gouvernements français et allemand veulent promouvoir les solutions européennes de confiance en matière de, ce qui va dans le bon sens. Toutefois, qu'en est-il de la traduction législative du rapport de notre collègue député Raphaël Gauvain, que le Gouvernement a annoncé à plusieurs reprises ? Qu'en est-il de la réforme de la loi de blocage, promise depuis plusieurs années ? Qu'en est-il de l'extension du règlement général européen Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous éclairer sur les intentions du Gouvernement sur ces points dans les dix-huit mois à venir ? Le Cyberscore que vise à instaurer cette proposition de loi permettra aux entreprises utilisant des solutions « grand public » d'être mieux informées. cela ne résout pas tous les problèmes auxquels nos entreprises doivent faire face quant à la sécurisation de leurs données. Monsieur le secrétaire d'État, malgré notre réel désaccord de ce matin et, je dois le dire, notre réel mécontentement sur le fond et sur la forme, nous sommes bien évidemment disposés à travailler avec vous sur ces sujets stratégiques pour notre économie et notre pays.

il est important de commencer à agir. J'entends bien que cette proposition de loi est incomplète et imparfaite, mais elle a le mérite de commencer à cadrer un certain nombre de sujets

La sécurité de ces données est essentielle ; il est de notre rôle de l'assurer. Malheureusement, la prise de conscience de l'importance de cette sécurité est loin d'être généralisée chez nos concitoyens. Finalement, les mesures à prendre en matière de cybersécurité recouvrent le même champ que celles qui sont préconisées actuellement en matière de sécurité sanitaire : mise en oeuvre de barrières, de restrictions, ou encore nettoyage systématique ...

La période de confinement que nous venons de traverser et le développement du télétravail interrogent sur cette conscience et sur la protection que nous proposons aux usagers. Ce fut réellement l'occasion d'une prise de conscience sur la fiabilité de ces différents logiciels. À ce stade, aucune disposition ne garantit l'information du consommateur quant à la sécurité informatique de la solution numérique utilisée. C'est l'objet principal de cette proposition de loi, portée par notre collègue Laurent Lafon. Afin que les consommateurs prennent davantage en compte les impératifs liés à la cybersécurité,

La mise en place de cette forme de Nutriscore numérique, également appelée Cyberscore, doit impérativement être simple, avec une information immédiate.

l'Union européenne doit également agir en construisant une nouvelle stratégie de cybersécurité d'ici à la fin de l'année 2020. Monsieur le secrétaire d'État, pourriez-vous nous éclairer sur ces engagements,

le numérique est décidément à l'honneur au Sénat : le 19 février dernier, nous adoptions à l'unanimité la proposition de loi de notre présidente Sophie Primas visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace- la liberté de choix des utilisateurs d'équipements terminaux et l'interopérabilité des services de communication au public en ligne étaient alors des points cardinaux de ce texte. Le 24 juin dernier, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable adoptait le rapport d'information de Guillaume Chevrollier et de Jean-Michel Houllegatte sur l'empreinte environnementale du numérique, après les six mois de travaux de la mission d'information que j'ai eu l'honneur de présider. Le Sénat n'a pas attendu la crise sanitaire pour se pencher sur les nouveaux enjeux du numérique. Force est de reconnaître que nous avons été bien inspirés. Disons-le simplement : les données, qui seront la matière première stratégique du XXI siècle, ne sont pas encore traitées avec la rigueur qu'il conviendrait de leur réserver. Les données informatiques ne doivent pas être confondues avec de l'information. Qu'il s'agisse de la gestion de volumes exponentiels, de la protection contre des utilisateurs malveillants ou encore du risque de manipulation, nous n'avons pas encore déterminé de politique publique idoine. Faut-il légiférer ? Que peut-on espérer du cadre communautaire actuel ? Doit-on attendre le futur, qui doit permettre, à terme, de définir un cadre de certification européen ? Toutes les questions que pose le développement exponentiel des usages ne trouveront pas de réponse aujourd'hui. Pourtant, cette proposition de loi s'attaque et, je le crois, répond à un chantier essentiel, celui de l'information du public sur la sécurité de l'information qu'il transmet aux plateformes numériques. Je citerai deux chiffres pour nous convaincre de l'importance du sujet

Aussi, comme le souligne le rapport de notre collègue Anne-Catherine Loisier, que je salue pour la pertinence de ses travaux, si les consommateurs sont protégés, en tant que personnes physiques, par le règlement général de protection des données adopté à l'échelon européen en 2016, ce dernier n'impose cependant pas d'informer sur la cybersécurité des solutions proposées par un prestataire de solutions numériques. Autrement dit, si le droit européen de la cybersécurité prévoit, à terme, des certifications harmonisées de cybersécurité, une telle certification reste, à ce jour, une démarche volontaire de l'entreprise concernée. L'article 1 de cette proposition de loi, qui oblige les plateformes numériques à fournir aux consommateurs un diagnostic de cybersécurité, afin de mieux

Je souscris au fait qu'il faille élargir le champ d'application du dispositif à tout fournisseur de services de communication au public en ligne. Je souscris également à la proposition de substituer un arrêté au décret définissant les indicateurs.

Désormais, seuls les indicateurs et la durée de validité devraient être fixés par arrêté. La rédaction actuelle de l'article 1 me semble donc cohérente, même si j'ai cru comprendre qu'elle pouvait encore évoluer d'ici à la fin de notre examen, notamment pour renforcer la cybersécurité des entreprises utilisatrices.

si elle inclut des objectifs particuliers. Les impératifs de cybersécurité ne concernant pas tous les marchés publics, cet ajout n'est peut-être pas indispensable. vous l'aurez compris, dans sa rédaction actuelle, et compte tenu des évolutions possibles que peut connaître ce texte en séance, notre groupe votera pour cette proposition de loi. La discussion

Ce travail a été poursuivi dans le cadre d'une commission d'enquête sur la souveraineté numérique que j'ai eu l'honneur de présider, laquelle s'est notamment appuyée sur le rapport de Gérard Longuet, dont je veux également saluer la contribution.

vise à modifier la rédaction de l'article 1, en rendant obligatoire pour les principaux opérateurs de plateformes en ligne la communication auprès de leurs utilisateurs d'un diagnostic de cybersécurité. Le Gouvernement propose ainsi de recentrer le dispositif sur les principaux opérateurs de plateformes en ligne, mentionnés à l'article L. 111-7-1 du code de la consommation.

En conséquence, il n'est pas nécessaire de prévoir, à l'article 1, qu'un décret fixe un seuil pour définir le champ d'application du dispositif, qui sera en effet celui de l'article L. 111-7-1 du code de la consommation. Plus simplement, nous cherchons à rendre le Cyberscore obligatoire pour les plus grandes plateformes les plus utilisées,

la notion d'opérateur de plateforme en ligne au sens du code de la consommation. Je rappelle que cette notion ne renvoie qu'aux services dont l'activité consiste en un référencement de produits en ligne ou en une mise en relation de personnes en vue de réaliser des échanges.

sans quoi, je le répète, des services initialement visés par la proposition de loi de notre collègue Lafon, comme les services de visioconférence en ligne, risqueraient d'être exclus du Cyberscore. Je comprends que le Gouvernement ne soit pas tout à fait en accord avec notre proposition de rédaction, mais, comme je l'ai dit, nous sommes disposés à retravailler ce dispositif ultérieurement. d'une contre-proposition satisfaisante, je vous propose donc de maintenir ce sous-amendement. En ce qui concerne le sous-amendement de M. Lafon, la commission n'a pas eu le temps matériel de se prononcer,

nous avons proposé- tel est l'objet de l'amendement n° 4 -que les modalités de présentation du diagnostic soient précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés du numérique et de la consommation. Il nous semble que la rédaction proposée par le Gouvernement permet d'atteindre l'objectif visé par le sous-amendement ; c'est dans cet esprit, avec la volonté d'afficher une signalétique claire, largement visible et probablement appuyée sur un système coloriel, qu'est rédigé l'amendement du Gouvernement, qui tend à renvoyer la définition de ces critères au niveau réglementaire,

Or, à la différence d'un critère comme celui du développement durable, qui est susceptible de concerner tous les marchés, le critère de la cybersécurité ne saurait porter que sur les achats de prestations informatiques. Le principe fondamental d'égalité devant la commande publique, qui impose de ne formuler d'exigence en termes d'expression des besoins, de critères de choix et de clauses d'exécution qu'en lien avec l'objet du marché, serait totalement bafoué. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement vous propose la suppression de l'article 2. l'avis de la commission ?

vote. Bien entendu, je voterai ce texte, que j'ai d'ailleurs souhaité cosigner, sur l'initiative de notre collègue Laurent Lafon, que je félicite, tout comme Mme la rapporteure Anne-Catherine

une réforme beaucoup plus structurelle que nous pourrons définitivement assurer, dans le cyberespace, la protection du consommateur et des données des citoyens et des

; la communication avec les utilisateurs en aurait largement pâti. Nous regrettons en particulier, dans cet amendement n° 4 du Gouvernement, l'abandon de l'obligation d'une évaluation des plateformes par une autorité administrative indépendante

au Parlement français dans son ensemble de s'approprier ces problématiques liées au numérique dans toutes leurs dimensions, sociales, sociétales, économiques, etc. Cette proposition reste tout à fait d'actualité ; je ne me résous pas, pour

Primas : plus nous prenons du retard, plus nous nous mettons en difficulté sur une question essentielle, la souveraineté numérique. Et lorsque l'on évoque cette question, il faut parler aussi d'industrie. Nous avons eu tout un débat, l'an dernier, sur la 5G.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la dotation d'équipement des territoires ruraux constitue, vous le savez, une dotation essentielle pour les communes et leurs groupements. Elle l'est plus que jamais, pour plusieurs raisons. La première raison, ce sont les baisses successives de la dotation globale de fonctionnement, la DGF, durant le dernier quinquennat ont représenté plus de 11 milliards d'euros, soit une diminution de 20 %, entraînant une réduction des capacités d'investissement des communes. J'ajoute que, malgré une stabilisation globale de l'enveloppe depuis le début de ce quinquennat, la baisse se poursuit pour certaines communes, puisque, dans le département dont je suis élu, plus de 300 communes ont connu une diminution de DGF entre 2017 et 2020.

qui a privé de nombreuses communes de précieux concours. Je le rappelle, ce dispositif permettait de financer principalement des petits projets de communes rurales, avec une très grande souplesse.

Lors de sa suppression en 2017, le Gouvernement avait annoncé dans un premier temps qu'une nouvelle dotation serait créée. Il n'en a rien été. Il s'est même opposé au dispositif adopté par le Sénat sur mon initiative, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018, qui prévoyait les mêmes avantages que la réserve parlementaire. Le Gouvernement a ensuite indiqué que la suppression de la réserve parlementaire serait compensée par une augmentation de la DETR. Il n'en a rien été non plus, puisque seuls 50 millions sur 150 millions d'euros que représentait la réserve parlementaire ont été réaffectés à la DETR. Dans certains départements, les effets n'en ont pas été ressentis. Ainsi, le montant de la DETR dans l'Eure a même connu une baisse entre 2017 et 2018. C'est dire que la DETR est devenue, dans de nombreux cas, indispensable à la réalisation et à la faisabilité d'un projet. La décision du préfet d'octroyer, ou non, cette subvention conditionne ainsi dans la plupart des cas le sort d'un projet. Son attribution doit donc être plus que jamais transparente et juste. Or, force est de constater que, malheureusement, la procédure d'attribution est, à plusieurs égards, insatisfaisante, et les choix des projets subventionnés peuvent, de ce fait, être l'objet de légitimes incompréhensions, voire de suspicions, de la part des élus. Si le cadre légal définit les critères d'éligibilité des collectivités locales à cette dotation, il a pu être observé dans certains cas l'introduction par le préfet dans le règlement départemental de critères qui excluent de fait et sans base légale des communes du bénéfice de la DETR.

Un autre élément particulièrement insatisfaisant est le rôle très limité de la commission des élus, tant par le cadre légal qu'en pratique, à tel point que la participation à ses réunions procure bien souvent le désagréable sentiment de participer à une structure totalement inutile. La loi prévoit que la commission des élus fixe les catégories d'opérations prioritaires à financer, ainsi que les taux de subventionnement plancher et plafond. Dans les faits, le préfet dispose de la capacité de retenir les projets de son choix sans être lié par les catégories retenues par la commission. J'ai pu ainsi observer des cas où le préfet a rejeté systématiquement les dossiers relevant d'un type d'opérations jugé pourtant prioritaire par la commission.

le préfet n'a pas l'obligation de rendre compte devant la commission de la liste des dossiers qu'il a sélectionnés et des critères appliqués pour choisir les projets à financer. Ces différentes limites conduisent à réduire la commission des élus à une instance d'enregistrement de choix unilatéraux du préfet, tout en donnant une apparence de concertation à cette procédure. L'objectif de cette proposition de loi vise donc à remédier à cette situation, sans toutefois remettre en cause le rôle décisionnaire du préfet. Elle tend à réaffirmer dans son article 1 le caractère exclusif de la loi dans la définition des critères d'éligibilité des collectivités locales à cette dotation. Aussi, les communes et leur groupement ne doivent pas pouvoir se voir opposer d'autres critères d'éligibilité à la DETR que ceux qui sont déjà prévus par la loi. L'article 2 tend à renforcer le rôle de la commission des élus et la transparence de la procédure d'attribution. Il convient ainsi de modifier le seuil de 100 000 euros précédemment évoqué, qui a pour effet de restreindre très fortement le rôle consultatif de la commission des élus. C'est pourquoi, dans la version initiale de ma proposition de loi, je proposais de supprimer ce seuil, afin que l'avis de la commission porte sur l'ensemble des dossiers. Le rapporteur vous exposera tout à l'heure les raisons qui l'ont conduit à une proposition de substitution, à savoir à un abaissement du seuil à 80 000 euros, plutôt qu'à une suppression pure et simple. J'ai bien sûr accepté cette solution de compromis.

Cette disposition permettra que la commission rende un avis éclairé, en connaissant les dossiers que le préfet compte subventionner comme ceux qu'il propose de rejeter. Il impose également que le préfet détaille pour chaque catégorie d'opérations les éléments sur lesquels il s'est fondé pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant. Il prévoit également une communication sur la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues. L'article 2 vise par ailleurs à inscrire dans le marbre de la loi l'obligation pour le préfet de respecter les catégories définies par la commission des élus. Enfin, l'article 3 de cette proposition de loi consacrait dans sa version initiale un « droit à l'erreur » au profit des communes et de leurs groupements dans le cadre de leur demande de subvention.

Ainsi, une omission, même minime, peut faire perdre dans certains cas le bénéfice d'une subvention à la collectivité locale. Le rapporteur a fait remarquer que cette disposition était déjà satisfaite par le cadre réglementaire, et il a en conséquence supprimé l'article 3 de ce texte. Il conviendrait donc que les préfets l'appliquent avec une plus grande rigueur ce dispositif. Nous sommes un certain nombre à pouvoir témoigner que ce n'est pas toujours le cas ! Mes chers collègues, je vous sais sensible à ces sujets, puisque notre Haute Assemblée a déjà adopté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018 les mesures prévues par ce texte visant à renforcer le rôle de la commission des élus et la transparence dans l'attribution de la DETR. Malheureusement, ces dispositions avaient été supprimées par l'Assemblée nationale, avec le soutien du Gouvernement, comme toujours ... J'espère que vous renouvellerez dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi, que votre commission des finances a adopté à l'unanimité, votre soutien à ces mesures, alors que nos communes, notamment celles de petite taille, sont encore plus dépendantes de ce dispositif à l'heure où leurs finances ont été fortement fragilisées par la crise sanitaire. J'espère également que le Gouvernement percevra enfin le bien-fondé de ce texte et donnera un avis favorable à son adoption au Sénat, puis à son examen et à son adoption l'Assemblée nationale. La parole

c'est un sujet bien connu des élus de la ruralité dont nous allons débattre maintenant : celui de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR. Il s'agit d'un outil financier de l'État très important pour des milliers de maires et d'élus des territoires ruraux, particulièrement dans les petites communes, car il soutient leurs projets d'investissement à hauteur de 1 milliard d'euros en 2020 ; plus de 20 000 projets ont pu en bénéficier. L'une des particularités de ce dispositif tient à la mise en place, dans chaque département, d'une commission composée d'élus locaux et de parlementaires, qui fixe les catégories d'opérations prioritaires, ainsi que les taux planchers et plafonds

C'est précisément sur le rôle de cette commission et la procédure d'attribution de la DETR que porte la proposition de loi de notre collègue Hervé Maurey. En effet, si dans l'immense majorité des départements les règles les règles d'attribution de la DETR et les prérogatives de la commission sont parfaitement respectées, dans le cadre de relations transparentes entre le préfet et la commission des élus, des cas de dysfonctionnement ont parfois été constatés. C'est pourquoi je partage C'est pourquoi je partage les préoccupations de notre collègue et l'esprit de sa proposition de loi, qui vise à éviter ces dysfonctionnements et à améliorer, là où c'est nécessaire, la transparence du processus. Toutefois, avec la commission, j'ai souhaité trouver un juste équilibre entre, d'une part, la nécessaire transparence des procédures et, d'autre part, le besoin de préserver réactivité et efficacité dans l'attribution des subventions : il y va de l'intérêt des collectivités et de leurs investissements. À cet effet, j'ai proposé, avec l'accord de son auteur, plusieurs amendements au texte initial que la commission a bien voulu adopter. L'article 1

tout projet porté par une commune au motif qu'elle ne se serait pas engagée dans une démarche de non-artificialisation des terres. Si l'appréciation de l'opportunité du financement des projets relève bien du préfet et, le cas échéant, de la commission,

Pour répondre à une question qui m'a été posée, il va de soi que cette disposition n'a aucunement pour effet de créer une obligation de subventionner automatiquement les projets présentés par une collectivité. L'article 2 comporte quant à lui diverses dispositions visant à renforcer le rôle de la commission DETR. Premièrement, il vise à enrichir l'information portée à la connaissance de la commission. à prévoir que toutes les demandes de DETR lui soient transmises, que celles-ci aient été retenues par le préfet ou non. Sur ce point, il me semble utile que les élus disposent de cette information. Aujourd'hui, leur vision se limite aux seules opérations retenues par le préfet. Je suis convaincu que cet effort de transparence est de nature à améliorer la qualité des travaux de la commission DETR et à éclairer son jugement, pour définir les opérations prioritaires et fixer les taux planchers et plafonds. Toutefois, la commission a voulu préciser le champ de cette nouvelle obligation d'information, qui ne concernerait évidemment que les dossiers complets et recevables. Par ailleurs, l'article 2 2 visait initialement à prévoir que la commission DETR soit saisie pour avis de l'ensemble des demandes de subvention, et non plus seulement des projets qui appellent une subvention supérieure à 100 000 euros. Je l'ai souligné en commission, je n'y suis personnellement pas favorable. Il me semble en effet que la suppression de tout seuil alourdirait considérablement la procédure et en allongerait les délais, au détriment de l'investissement des collectivités territoriales. Il faut, me semble-t-il, laisser aux préfets une certaine souplesse,

et en accord avec l'auteur de la proposition de loi, la commission des finances a adopté un amendement visant à abaisser de 100 000 euros à 80 000 euros le seuil au-delà duquel une saisine pour avis de la commission est requise.

Enfin, l'article 3 de la proposition de loi initiale visait à instaurer un « droit à l'erreur » pour les collectivités dans leur dossier de demande de subvention au titre des dotations de l'État. sous-tendait cet article 3 était simple : une commune ne doit pas pouvoir se voir refuser la subvention au seul motif que son dossier serait incomplet, sans même lui avoir laissé la possibilité de le compléter dans un délai raisonnable. Là encore, l'auteur de la proposition m'a fait part d'une situation locale tout à fait inadmissible, où une commune au dossier incomplet perdait toute chance de se voir octroyer la DETR. toutefois proposé à la commission de supprimer cet article. Cette suppression ne traduit en aucun cas une opposition de principe de la commission. Elle relève simplement que le droit à l'erreur est déjà garanti par les textes en vigueur. En effet le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction actuelle, dispose que dans le cas d'un dossier incomplet le préfet doit demander les pièces manquantes dans les trois mois

Pour terminer, monsieur le secrétaire d'État, je voudrais attirer votre attention sur deux difficultés rencontrées par les élus locaux et pour lesquelles des solutions pourraient être envisagées. La première concerne la date d'attribution des subventions DETR. Chaque début d'année, les élus attendent avec impatience la décision du préfet pour l'attribution ou non de la subvention DETR, car elle conditionne la plupart du temps la mise en oeuvre de leurs projets. Ils doivent souvent voter le budget de leur commune avant même de connaître la réponse, et par conséquent sans pouvoir inscrire les dépenses et recettes affectées à leur projet.

Deuxième difficulté, les crédits non consommés et qui n'ont pas été redéployés dans l'année en cours doivent être restitués et sont donc perdus pour le département. Or les raisons de cette sous-consommation sont la plupart du temps indépendantes de la bonne gestion des collectivités.

je me réjouis de me trouver parmi vous, pour la première fois au Sénat dans mes fonctions de secrétaire d'État chargé de la ruralité, pour examiner un texte relatif aux collectivités territoriales. Bien que je n'aie jamais siégé à la chambre haute, nous avons en partage, vous le savez, ce beau sujet de l'aménagement de l'espace rural. Et c'est bien de ruralité que nous allons discuter cette après-midi, en nous penchant sur la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR. Il s'agit d'ailleurs d'un sujet qui ne m'est pas totalement étranger, car, avant ma nomination au Gouvernement, j'étais justement corapporteur avec la députée Christine Pires Beaune, et sous la présidence de Jean-René Cazeneuve, président de la délégation aux collectivités territoriales de l'Assemblée nationale,

J'espère qu'elle pourra aboutir rapidement, en vue d'éventuelles propositions pour la seconde partie du projet de loi de finances. Les choses sont à mon sens bien parties. Les sénateurs Hervé Maurey et Bernard Delcros ont parfaitement décrit le caractère absolument essentiel de la DETR pour le financement des investissements dans les territoires ruraux. J'aimerais simplement revenir sur quelques points et vous faire part de mes réserves sur les articles du texte inscrit à l'ordre du jour. Je rappelle que la DETR, c'est d'abord une enveloppe de plus de 1 milliard d'euros de crédits : 1,046 milliard pour être précis. J'insiste un peu sur le chiffre, car, vous le savez tous, en 2014 la DETR s'élevait à environ 600 millions d'euros : aujourd'hui, c'est 60 % de plus. Vous avez d'ailleurs constaté que l'enveloppe est sanctuarisée dans le projet de loi de finances pour 2021, en dépit du fait que plusieurs milliards d'euros de crédits soient ouverts par ailleurs en faveur des territoires dans le plan de relance. Je crois que cette stabilité de la DETR, budget après budget, est un bon signal adressé aux 30 000 communes rurales de France : c'est la preuve que cette dotation est incontournable dans le paysage des finances locales et qu'elle le restera. C'est en tout cas mon souhait, et vous pouvez compter sur moi pour la défendre. La DETR, ce sont aussi des modalités de gestion particulières, adaptées aux besoins des communes rurales. Contrairement aux autres subventions d'investissement, la DETR est gérée à la fois de manière déconcentrée et décentralisée.

Ces priorités diffèrent d'un département à l'autre : ici, les élus demandent au préfet de faire un effort sur les routes ; là, sur les réseaux d'assainissement. Ce système permet que la DETR aille bien régler des questions locales qui se posent à certains endroits, mais pas partout. Les orientations fixées par l'État sont donc indicatives :, ce sont les élus locaux qui fixent les règles du jeu. Par ailleurs, elle contrôle l'utilisation des crédits en rendant un avis sur les subventions supérieures à 100 000 euros. Pourquoi ce seuil ? Tout simplement parce qu'il permet de concilier, comme l'a rappelé à l'instant M. le rapporteur, un travail efficace, rapide et raisonnable de la commission qui examine en moyenne 16 % des subventions, tout en contrôlant une grande part des crédits, soit 58 % des enveloppes budgétaires. C'est ce qu'à Bercy ou dans mes précédentes fonctions de rapporteur général j'aurais appelé un bon contrôle hiérarchisé de la dépense ! Bien entendu, ce n'est pas la commission, qui se réunit en moyenne deux fois par an, parfois trois, qui reçoit les dossiers, les instruit, les sélectionne et les valide. C'est le rôle de l'État, en l'occurrence du préfet. Des modifications significatives ont été mises en oeuvre depuis le début du quinquennat, afin de renforcer la transparence de la gestion de la DETR et de mieux associer les élus. Bon nombre d'entre elles ont

La commission a été élargie aux parlementaires du département : tous en sont membres quand il y a moins de cinq parlementaires, ce qui est le cas chez moi dans les Hautes-Alpes, où nous n'avons que deux députés et un sénateur. Le seuil d'avis a été abaissé de 150 000 euros à 100 000 euros, permettant de passer d'un examen de 42 % à 58 % des crédits aujourd'hui.

ainsi que les orientations qu'il entend retenir pour celle-ci pour l'année en cours. Je ne suis pas là pour accorder un satisfecit général sur la DETR, mais je crois que, dans l'immense majorité des départements, même s'il peut y avoir des exceptions, les élus font le constat que le système fonctionne

tout en profitant de la moindre erreur de parcours des communes pour leur refuser des subventions ... C'est un tableau très éloigné de la réalité que je connais. J'ai été maire pendant vingt-sept ans, membre de la commission DETR pendant le même nombre d'années, et je n'ai, en tout état de cause, jamais constaté la moindre entorse au dialogue républicain entre la préfecture et les maires sur ce sujet. Certes, il existe sans doute des exceptions. J'en prends acte, mais le ministère que je représente et le Gouvernement sont là pour étudier avec vous les difficultés qui pourraient remonter au niveau central. Mon message est donc simple : les évolutions récentes sont de vraies avancées. Il faut donc exploiter à plein la procédure existante et toutes les possibilités qu'elle offre. À l'inverse, les évolutions prévues dans la proposition de loi pourraient brouiller les rôles respectifs de l'État et de la commission et remettre en cause le point équilibre atteint aujourd'hui dans la plupart des départements. pourquoi le Gouvernement ne sera pas favorable aux deux articles de la proposition de loi. Je m'en explique. L'article 1 tend à prévoir que les communes et EPCI qui satisfont les conditions démographiques d'éligibilité à la DETR « ne peuvent se voir opposer aucun autre critère d'éligibilité à cette dotation ». Il faut s'entendre sur le sens de cette disposition : soit elle signifie que ni le préfet ni la commission n'ont le droit de fixer de cadre d'emploi à la DETR, ce qui est évidemment impossible, car les communes auraient une sorte de droit de tirage sur la elle signifie que la commission a seulement le droit de fixer des priorités des projets, mais pas des critères d'éligibilité des communes. Si c'est cette dernière interprétation qui prévaut, alors nous sommes d'accord, mais il s'agit déjà du droit applicable.

Quant à l'article 2, il vise à modifier la répartition des rôles entre le préfet et la commission, ainsi que les équilibres internes à la commission, en y intégrant jusqu'à six parlementaires, en portant à sa connaissance les projets déposés, mais refusés, en abaissant le seuil d'avis à 80 000 euros ou en demandant au préfet de justifier les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour faire ses choix. Je pense que cet article aurait des conséquences concrètes que les élus ne souhaitent pas, sans apporter de plus-value réelle au travail de la commission. Par exemple, introduire davantage de parlementaires dans la commission souvent à ce que la réunion compte davantage de députés et de sénateurs que de maires et de présidents d'EPCI, alors que c'est bien à eux que s'adresse la DETR. Je ne crois pas que les associations d'élus locaux, telles que l'Association des maires ruraux de France, l'AMRF, que je rencontre et consulte fréquemment, soient favorables à une telle proposition Autre exemple, je ne connais aucun maire rural qui demande que la commission ait connaissance du projet refusé, que le préfet aura peut-être tout simplement décidé de réserver pour l'exercice suivant, souvent en bonne intelligence avec l'élu local. J'insiste un peu sur ce point : il est normal et sain

Dernier exemple, l'abaissement du seuil à 80 000 euros conduirait les commissions à examiner 1 000 dossiers de plus par an, dont le démarrage serait donc conditionné à une réunion en bonne et due forme. C'est compréhensible pour les gros projets,

Je suis en revanche tout à fait ouvert à ce que les préfets fournissent aux commissions et aux parlementaires des informations générales sur les critères ayant permis de retenir les dossiers.

arrive devant la Haute Assemblée dans un contexte économique inquiétant pour l'avenir financier des collectivités. La crise sanitaire que nous connaissons, hélas, aggrave les difficultés que rencontrent déjà nos territoires ruraux. Plus que jamais, il est nécessaire d'ajuster le fonctionnement de la DETR aux réalités qui s'expriment sur le terrain. Cette dotation est le symbole du besoin constant et du devoir vigilant qui nous incombe, celui de repenser l'interaction entre l'État et les collectivités, de défendre ces dernières et de porter leur voix. En soutenant les investissements des communes et des intercommunalités, et à côté d'autres dotations, la DETR représente un enjeu financier de taille, contribuant au développement des territoires, à la relance de l'économie locale et à l'articulation des projets. Au demeurant, et malgré la montée en puissance de cette dotation, plusieurs acteurs relèvent son manque d'efficacité. Une vigilance accrue doit donc être portée à la dynamique des finances locales. À cet égard, cette proposition de loi est intéressante. Elle permet de rendre la procédure d'attribution de la DETR plus accessible et transparente. Elle conforte également son rôle de fixation des opérations prioritaires et de leur taux de subvention. L'abaissement du seuil au-delà duquel une saisine pour avis de la commission DETR est requise à 80 000 euros nous semble aller dans le bon sens. Cependant, d'autres améliorations nous paraissent envisageables. À titre personnel, je vis la ruralité au quotidien depuis 1994 : vingt-six années au cours desquelles j'ai endossé les responsabilités de maire, puis de président de communauté de communes. j'ai appris les difficultés du quotidien liées à l'éloignement géographique, à la désertification, à l'isolement parfois, mais surtout au manque de moyens financiers et humains. Aujourd'hui encore, il existe un différentiel entre les crédits disponibles et les crédits consommés, souvent dû au manque d'ingénierie de moyens des petites collectivités. Une analyse plus complète serait nécessaire sur ce point, car il est souvent impossible de prendre en charge la DETR les dépenses des études préalables, pourtant indispensables. Sur ce point, une information régulière du préfet à destination de la commission DETR sur les crédits restant disponibles serait souhaitable. Enfin, comme il appartient à la commission DETR de fixer les catégories d'opérations prioritaires, nous souhaiterions que l'écoconditionnalité d'un projet puisse être retenue pour allouer une fraction supplémentaire de dotation. À titre d'exemple, en Corse ou dans d'autres régions, les projets qui favoriseraient l'utilisation des ressources locales, comme le bois, pourraient se voir attribuer un pourcentage de subvention supplémentaire.

La valorisation des ressources locales est à l'heure actuelle au coeur des recherches et des expérimentations sur les leviers du développement économique dans les territoires ruraux. Ainsi, nous pourrions soutenir un modèle de développement basé sur une utilisation durable de l'environnement, les territoires sont porteurs de démarches de valorisation des ressources locales. Je conclurai en rappelant que la diversité de nos territoires et les contraintes de la ruralité sont constitutives de notre identité profonde. Nous devons y consacrer une attention particulière eu égard à l'égalité des chances, parfois mise à mal dans nos territoires. Je connais le formidable potentiel de la ruralité, mais aussi son extrême fragilité. Au sein de mon groupe, je serai donc porte-parole de ces petites communes. À cet égard, le texte que nous examinons est vertueux, car il permet d'avancer vers une efficacité accrue de l'attribution de la DETR. Pour toutes ces raisons, les sénateurs du groupe Écologiste-Solidarité et Territoires y sont favorables. La parole

C'est un levier indispensable dans les projets soutenus par les élus, comme nous le mesurons lors de chacun de nos déplacements ou inaugurations dans les communes de nos départements. Depuis 2011 les montants ouverts en loi de finances ont connu une augmentation très significative : entre 2011 et 2014, le montant ouvert était d'environ 616 millions d'euros en 2015 et en 2016, il a atteint 816 millions d'euros ; en 2017, il a été porté à 996 millions d'euros, puis à plus d'un milliard d'euros depuis 2018. La DETR obéit aussi à une logique de décentralisation, et tant mieux. En effet, la décision d'attribuer les subventions relève du préfet de département, dans le cadre fixé à l'échelon de chaque département par une commission d'élus. D'importantes avancées ont été récemment apportées dans le fonctionnement de la commission, afin de renforcer l'information des élus et la transparence des travaux. Depuis 2018 par exemple, les membres de la commission sont destinataires avant chaque réunion d'une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour, du jour, note également communiquée à l'ensemble des parlementaires du département, lesquels sont d'ailleurs membres de la commission depuis 2017. L'objet de cette proposition de loi est de renforcer le rôle de la commission, de fluidifier et de compléter le niveau d'information des membres de la commission, de faire en sorte qu'il y ait davantage de transparence entre les élus et le préfet. Sur le principe, nous ne pouvons qu'en rejoindre l'esprit, mais, concrètement, ce texte pose quelques difficultés. en termes de philosophie, avec cette proposition de loi, c'est-à-dire sous le sceau du législateur, le principe est de rigidifier davantage les règles fixées pour la DETR. Si des invraisemblances existent dans certains départements, cela peut très bien être clarifié par circulaires aux préfets, aux préfets, qui sont tenus de respecter les priorités définies dans les commissions départementales. Dans le détail, l'article 1 du texte inscrit dans la loi que les communes et EPCI qui satisfont les conditions démographiques d'éligibilité à la DETR « ne peuvent se voir opposer aucun autre critère d'éligibilité à cette dotation. Du coup, ne doit-on pas s'interroger sur le rôle et la légitimité de la commission ? L'impossibilité d'écarter tout type de projet qui ne serait pas défini collégialement dans cette instance pourrait être considérée comme une restriction des pouvoirs de la commission, et donc un retour en arrière quant au caractère décentralisé de ses compétences. L'article 2 prévoyait initialement de transmettre la liste de toutes les opérations faisant l'objet d'une demande de subvention à la commission. Un problème se pose : il n'est pas certain que le maire soit très enthousiaste à l'idée de soumettre son projet à l'ensemble de la commission d'élus

Toujours à l'article 2, il était question de saisir pour avis la commission de l'ensemble des projets, quel que soit leur montant. Cela paraissait infaisable et de nature à alourdir techniquement la procédure d'attribution. L'abaissement du seuil de consultation à 80 000 euros va également dans le bon sens, mais il convient de veiller à ne pas engorger la commission.

Par ailleurs, l'article 2 institue une obligation pour le préfet de motiver des décisions d'acceptation et de refus. Là encore, c'est un bon outil de lisibilité de l'information pour la commission.

cette proposition de loi est trop coercitive et trop centralisatrice. L'examen de cette dernière permet publiquement de témoigner des difficultés et interrogations qui se posent au cas par cas dans certaines commissions, et tel est le rôle du Sénat. Nous attendons donc du Gouvernement des réponses à ces difficultés, mais nous ne sommes pas certains que ces réponses soient de nature législative. Le groupe Rassemblement

c'est avec beaucoup d'émotion que je m'exprime aujourd'hui à la tribune du Sénat, pour la première fois depuis mon élection, le 27 septembre dernier. Je tiens à remercier de nouveau les élus de mon département, l'Hérault, qui m'ont ouvert les portes de la Haute Assemblée. J'ai également une pensée pour les Pérétoises et les Pérétois, les quelque 1 000 habitants de la commune de Péret, dont j'ai été le maire pendant trente-sept ans, de 1983 à 2020. Cette expérience au plus près des problèmes concrets de mes concitoyens a été déterminante dans mon parcours

Ces responsabilités m'ont donné le goût des chiffres, des finances locales et une connaissance des contraintes budgétaires pesant sur les communes, plus particulièrement dans les territoires ruraux. Voilà pourquoi, mes chers collègues, j'ai souhaité rejoindre la commission des finances à mon arrivée au Sénat.

L'article 2 vise, notamment, à améliorer la transparence de la procédure d'attribution. Il prévoit, d'une part, que l'ensemble des dossiers déposés par les collectivités locales soit porté à la connaissance des élus, quel que soit le montant de subvention demandé, et, d'autre part, que la commission rende un avis sur tous ces dossiers. cet article également, le préfet doit tenir compte des priorités fixées par la commission pour définir la liste des opérations à subventionner et justifier ses choix et les critères de sélection ou de rejet.

Comment, dans ce contexte, assurer l'attractivité de nos territoires ruraux sans octroyer davantage de financements pour soutenir les plus petites communes dans leurs projets les plus modestes ? Ces dépenses participent à la lutte contre la désertification rurale et sont à ce titre primordiales, davantage encore dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons. Le groupe RDSE est très attaché à tout ce qui peut contribuer à résoudre cette problématique. Avant de conclure, je précise que d'autres améliorations me sembleraient utiles. Il s'agit, par exemple, de prendre en compte non pas la population, mais uniquement le nombre de communes pour la répartition de la dotation par arrondissement. J'avais déposé un amendement en ce sens, que j'ai finalement décidé de retirer, une telle évolution relevant selon moi davantage du domaine réglementaire, voire du niveau de la circulaire.

Cela reflète souvent l'état des relations entre l'exécutif et les élus locaux avec un gouvernement qui a tendance à faire des économies sur le dos des collectivités, notamment à l'occasion de sa gestion actuelle de la crise. La DETR est intéressante puisqu'elle est liée à une commission instituée dans chaque département, composée d'élus locaux et de parlementaires. Comme les associations d'élus, mon groupe regrette que seule la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL)

Nous saluons le travail effectué dans le cadre de cette proposition de loi pour renforcer la transparence et la proximité de cette commission. Les priorités fixées par la commission demeurent évidemment dans un cadre législatif national, afin qu'il y ait une égalité des collectivités devant la loi

saisine permettra à la commission de se prononcer sur les projets représentant près de deux tiers des crédits octroyés. Une meilleure communication et une plus grande transparence de la part du préfet sur les motivations à l'origine de dossiers acceptés ou refusés, avec un détail des critères utilisés, complèteront ces avancées.

Au-delà de ces propositions, l'examen d'un texte relatif à la DETR permet de nous rendre compte que la notion de ruralité est à géométrie variable. En raison du manque de clarté du périmètre de la ruralité, ruralité, la DETR est attribuée en partie à des collectivités non rurales, c'est-à-dire de plus de 2 000 habitants, car 67 % des communes de plus de 3 500 habitants perçoivent cette subvention. Alors que l'Insee a récemment mis en place un groupe de travail chargé de proposer une définition statistique des espaces ruraux, nous estimons que le Parlement devrait être mieux informé de la répartition de la DETR en fonction du type de collectivité, mais également de sa capacité financière. Une mission d'information a été créée à l'Assemblée nationale, mais ses travaux ont été perturbés par la crise- n'y voyez pas un élément de polémique, c'est une réalité factuelle,

et de la dotation de développement rural (DDR). Il s'agit de la dotation de soutien aux investissements des collectivités locales la plus importante en volume. Depuis sa création, les montants ouverts en loi de finances ont connu une augmentation très significative, dans un contexte

La gestion de la DETR obéit à une logique de déconcentration et de décentralisation. La décision d'attribution des subventions relève du préfet de département, dans le cadre fixé à l'échelon de chaque département par une commission d'élus. Cette commission détermine à la fois les catégories d'opérations prioritaires

Depuis 2018, les membres de la commission sont destinataires avant chaque réunion d'une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'heure du jour, celle-ci étant également communiquée à l'ensemble des parlementaires du département. En 2018, le seuil au-delà duquel la commission rend un avis a été abaissé de 150 000 à 100 000 euros, ce qui a permis aux commissaires d'examiner cette année près de 2 900 dossiers- « seulement » ... Cette articulation entre la déconcentration des crédits et une logique de décentralisation permet à la DETR d'apporter un soutien décisif aux priorités qui sont celles du monde rural, en adaptant les stratégies de programmation aux besoins locaux. La DETR a exercé en 2018 un véritable effet de levier en contribuant à réaliser près de 4 milliards d'euros d'investissements dans ces territoires. Elle joue un rôle très complémentaire de la DSIL en finançant des projets de proximité, en particulier ceux qui sont soutenus par les petites communes pour des montants parfois très modestes. Les règles de gestion de la DETR permettent d'adapter la programmation aux besoins du département, s'agissant par exemple des priorités ou des taux de subvention. Certaines priorités communes aux territoires ruraux ont fait l'objet d'efforts spécifiques transition écologique, école et gendarmerie, rénovation thermique et aide au maintien des services publics, dont on connaît l'importance dans ces zones. Néanmoins, je partage les préoccupations de l'auteur de la proposition de loi. Si les règles d'octroi de la DETR sont respectées dans la très grande dans la très grande majorité des cas- je veux bien le reconnaître -, et si les relations entre la commission d'élus, le préfet et les services de l'État ne posent pas de difficultés majeures, des dysfonctionnements ont pu être constatés localement. J'en ai moi-même été témoin. Certaines de ces difficultés

L'article 1 concerne les critères d'éligibilité des communes à la DETR, qui sont définis par la loi. Dans un département, nous avons pu constater que le règlement départemental établi sur proposition du préfet excluait par principe certaines communes, pourtant éligibles au regard des critères déterminés par la loi. La rédaction du code général des collectivités territoriales qui résulterait de cet article 1 permettrait de lever toute ambiguïté sur ce point. L'article 2 comporte plusieurs dispositions qui tendent à renforcer le rôle de la commission, grâce à une transparence et une information accrues. défaut, le rôle de la commission deviendrait théorique. Cet article enrichit l'information apportée à la commission, qui aura connaissance de tous les dossiers déposés, qu'ils aient été ou non retenus par le préfet. J'ai bien entendu que vous n'y étiez pas favorable, Néanmoins, je pense que c'est utile, afin que la commission puisse définir ses priorités et les taux de subvention. L'article 2 prévoit également que la commission soit saisie pour avis de tous les dossiers de demande de subvention, et non pas seulement de ceux pour lesquels le préfet propose une subvention supérieure à 100 000 euros. Je me suis interrogée sur ce point : cette mesure me semble compliquée et risque d'alourdir considérablement la procédure

Cela se fait déjà dans de nombreux départements, notamment le mien, mais manifestement pas partout. L'article 3 visait à instaurer un droit à l'erreur pour les collectivités territoriales pour ce qui concerne la constitution et le dépôt de leur dossier de demande de subvention au titre des dotations de l'État. Or cette disposition est satisfaite par le droit

Ce texte à un sens tout particulier, puisqu'il a pour ambition de rendre cette procédure plus transparente et accessible, dans un seul but : l'efficacité. C'est pourquoi je tiens personnellement à saluer Hervé Maurey pour cette initiative Pour nos élus ruraux, pour nos concitoyens, une telle proposition de loi honore également le rôle du Sénat. Car nous, sénatrices et sénateurs, sommes des acteurs de terrain, proches des élus locaux et de leurs réalités. Notre rôle, notamment, est justement là : les défendre. En effet, trop souvent, les communes rurales et leurs habitants sont oubliés, au bénéfice des grandes villes et de leurs visibles et médiatiques « grands projets ». Le texte conforte le rôle des élus locaux, lequel consiste à fixer les catégories prioritaires, ainsi que les taux de subvention applicables. Cette disposition permet de défendre les petites communes qui rencontrent toutes, nous le savons, de croissantes difficultés financières. Cette proposition de loi permet, enfin, d'améliorer et de renforcer le rôle des commissions d'élus car, aujourd'hui, le rôle consultatif de ces commissions est limité, voire- osons le dire -carrément bridé.

de loi, je le répète, va dans le bon sens. Elle soutient les territoires ruraux et le juste octroi de leurs dotations. J'ai personnellement cosigné un certain nombre d'amendements visant à appuyer et à renforcer les aides aux élus des petites communes, qui en ont tant besoin. Soyons ambitieux pour nos petites communes. Aujourd'hui et maintenant, tous ensemble, préservons leurs moyens financiers. Permettons-leur de participer pleinement à cette grande relance économique si nécessaire à nos territoires. Envoyons à nos élus, aux maires de France un signal fort, donnons-leur des moyens ! Depuis le début de la crise sanitaire et de la crise économique, les communes, les intercommunalités et nos élus apportent, quant à eux, des réponses concrètes. Ils doivent répondre au quotidien aux besoins des habitants et des entreprises locales.

Évidemment, dans l'état actuel, celle-ci n'est pas non plus informée de l'ensemble des demandes formulées. Bref, il n'y a que peu de transparence, voire aucune, sur les dossiers en amont, donnant une effectivité toute relative à cette consultation des élus qui ne se prononcent ainsi que sur une infime partie des besoins de nos communes ou EPCI. Fruit de la fusion de la dotation de développement rural et de la dotation globale d'équipement des communes en 2011, et, dans une certaine mesure, de feu la réserve parlementaire en 2018, la DETR doit répondre aux besoins d'équipement des territoires ruraux.

Il nous avait alors été dit que ces sommes seraient reversées vers la DETR, puis ciblées en direction des petites communes. Mais force est de constater que, sur les deux années écoulées, le compte n'y est pas. pas. Dans mon département, qui compte 800 communes, dont presque 600 de moins de 500 habitants, le mot « rural » est dominant, et les besoins en investissements structurants, même petits, sont légion. Résultat, avec le relèvement systématique du plafond- de ce fait, les petits dossiers échappent à la vigilance de la commission personne ne peut plus mesurer l'étendue des besoins correspondants. C'est ainsi que les conditions d'attribution ont été très régulièrement évoquées par mes interlocuteurs durant cette campagne électorale. Pour l'année 2020, l'appel à projets a été lancé par circulaire du 7 janvier 2020, avec un dépôt limite

que l'augmentation des dépenses immédiates relatives à la protection de la population, mais aussi la baisse induite des recettes fiscales. De plus, 30 millions d'euros sont globalement prélevés sur la fiscalité propre de mon département au titre de la suppression de la taxe d'habitation, pour ne citer qu'un exemple. Ces deux facteurs conjugués vont représenter un coût très important pour les finances locales. Par ailleurs, l'immobilisation des entreprises durant le confinement et la difficile reprise de l'activité ont perturbé fortement l'investissement public, dont la DETR est un véritable levier. Aussi, compte tenu de la baisse continue des dotations, et parce qu'elle souffre d'un carcan certain, la DETR nécessite une adaptation à la réalité. Il va falloir nécessairement assouplir son fonctionnement. Je salue donc les dispositions de la proposition de loi et les améliorations apportées par le rapporteur, comme la fin des critères additifs départementaux excluant du bénéfice de la DETR, la communication de tous les dossiers déposés, une information plus complète et la baisse du seuil. Je soutiens également une partie des amendements qui ont été proposés. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la chaîne d'exécution ayant pris beaucoup de retard- dans certains cas, il n'y a même pas de commencement de travaux -, il paraît nécessaire de revoir la durée de validité de la demande de subvention, tout comme les délais réglementaires de commencement et d'achèvement de l'opération- ceux-ci pourraient être allongés d'un exercice supplémentaire. Pourquoi ne pas envisager également le déblocage des aides publiques tout au long de l'année, dès lors qu'un projet d'investissement a été déclaré éligible ? La relance des territoires par le biais des commandes publiques aux entreprises du BTP passera par une DETR plus souple, inclusive, argumentée et motivée, aussi bien lors de l'octroi que lors du refus,

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, il est un risque que nous prenons souvent en tant que parlementaires lorsque nous abordons des sujets aussi cruciaux pour les élus locaux que la décentralisation et l'aménagement du territoire : accorder plus d'importance à la théorie qu'à la pratique, en fait perdre pied avec le terrain.

Ce texte soulève des problèmes techniques, mais y apporte des solutions politiques, au bon sens du terme, car il pose la question de la prise de décision dans le cadre très précis de la DETR. La DETR- faut-il encore le rappeler ? -constitue un élément structurant pour nos politiques d'aménagement du territoire, avec une enveloppe d'un milliard d'euros pour les territoires. Elle participe à la cohésion de la Nation en opérant des transferts au bénéfice de la ruralité et des petites communes. Mais si nous sommes tous très attachés à ce dispositif vital pour le développement de nos territoires, nous n'en sommes pas moins regardants et exigeants quant à sa mise en oeuvre concrète. Le texte dont il est aujourd'hui question apporte à cet égard des solutions pragmatiques. La première de ces solutions concerne le champ d'application du dispositif. À l'heure actuelle, de nombreuses communes qui répondent à un appel à DETR se voient opposer un critère d'inéligibilité qui les prive de ce levier de développement. Pour répondre à ce problème, l'article 1 consacre le principe d'universalité de la DETR en modifiant directement l'article du code général des collectivités territoriales qui institue la DETR. Il vise ainsi à clarifier la loi. L'article 2 apporte des solutions techniques aux problèmes rencontrés sur le terrain dans la procédure d'octroi de la DETR. La méthode retenue me semble bonne : réinjecter de la décision politique dans les procédures administratives. Je pense bien sûr au seuil des 100 000 euros. Ce seuil marque de façon symbolique, mais assez symptomatique, le point de bascule entre décision administrative et décision politique : en deçà, c'est l'apanage du préfet ; au-dessus, la décision est partagée avec les élus.

C'est aux élus des territoires de prendre les décisions, de concerter, et de représenter les intérêts parfois divergents, souvent convergents, des différents acteurs des territoires. C'est dans la même logique que nous abordons les autres mesures de cette proposition de loi, telles que les obligations faites aux préfets de respecter les orientations prises par la commission des élus et de rendre compte des raisons pour lesquelles ils choisissent de rejeter des demandes de subvention. Je pense aussi à la meilleure représentation des parlementaires au sein de la commission DETR. Les dispositions contenues dans cette proposition de loi vont dans le bon sens, mais je présenterai un amendement, proposé par mon collègue Jean-Pierre Decool, qui vise à élargir cette mesure aux départements qui comptent au moins quinze parlementaires. Vous l'aurez compris, le groupe Les Indépendants - République et Territoires accueille très favorablement cette proposition de loi. Celle-ci permettra de matérialiser de façon concrète le souhait formulé par nombre de nos concitoyens : redonner du pouvoir au local et rapprocher la décision du terrain. Il s'agit non pas de jouer de façon simpliste le politique contre l'administration, mais bien de redynamiser la décision politique à l'échelon local. La

et du rapporteur de cette proposition de loi réformant la procédure d'octroi de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Comme ils l'ont rappelé, la DETR vise à un juste équilibre entre transparence et efficacité des procédures. Elle me semble participer à notre souci commun que la décentralisation au quotidien fonctionne à partir des projets des territoires, et non dans un cadre contraint qui en limiterait le champ des possibles. C'est donc une bonne chose que toutes les demandes de dossiers, complets et recevables, soient connues par la commission départementale, car cela permettra de mieux identifier les projets sur le territoire et d'adapter, si besoin, les catégories d'opérations prioritaires retenues par la commission départementale. Abaisser à 80 000 euros le seuil de subvention au-delà duquel la saisine est requise va également dans le bon sens, en ouvrant la concertation sur un plus grand nombre de dossiers. Il sera Il sera intéressant de faire une évaluation de cette mesure, afin de s'assurer de la pertinence du maintien de ce seuil ou de son abaissement à 50 000 euros dans les années à venir. Enfin, le rappel qu'aucun autre critère que ceux qui sont fixés par la loi ne peut justifier une inéligibilité conforte l'importance que nous accordons au respect du projet, tel qu'il est librement élaboré par les collectivités qui le présentent. la DETR est une dotation essentielle pour les territoires ruraux, et elle doit être au plus près des besoins des élus. Elle est aussi un outil important au service de la relance territoriale voulue par le Gouvernement. De ce point de vue, on peut regretter que le milliard d'euros supplémentaires affecté à la DSIL dans le plan de relance ne soit pas alloué à la DETR, au moins pour une part cela aurait permis de financer plus rapidement les projets et de favoriser la concertation entre l'État et les collectivités territoriales sur le développement des territoires. J'ajoute que, compte tenu des priorités retenues par l'État pour le fléchage de la DSIL supplémentaire, en déterminant les opérations éligibles, les plus petites collectivités sont de fait écartées. Les financements accordés au titre de la DSIL seront concentrés sur les plus grandes collectivités et, par nature, ne produiront pas d'effets sur l'économie réelle avant plusieurs mois. 60 % de l'investissement public national est réalisé par les communes : toutes y contribuent à proportion de leur taille. C'est souligner et redire leur importance dans la réussite de la politique de relance engagée par l'État.

Le plan de relance n'a pas considéré les communes comme des acteurs économiques dont il convenait de soutenir l'équilibre financier dans une période difficile, à la différence du parti pris pour le secteur privé. Ce choix a pour conséquence que le bloc communal reconstituera d'abord sa capacité d'autofinancement, en privilégiant l'épargne de précaution sur l'investissement. Cela conduit mécaniquement, dès cette année, à une baisse durable des capacités d'investissement du bloc communal dans un contexte de recentralisation progressive de ses recettes, transformées à marche forcée en dotations de l'État. L'expérience nous montre que ce mécanisme a toujours conduit à une diminution des ressources locales. C'est pourquoi le texte que nous examinons cet après-midi, dans le contexte financier que je viens de rappeler, s'inscrit en parfaite cohérence avec les propositions de loi étudiées par le Sénat cette semaine pour le plein exercice des libertés locales.

coeur de notre vocabulaire d'élus un sigle est incontournable : DETR. Tous les maires, conseillers départementaux et régionaux, et parlementaires le connaissent. Dans le contexte financier qui a vu les dotations globales de fonctionnement des communes des communes fondre comme neige au soleil entre 2014 et 2017, avant de se stabiliser à un niveau médiocre, la désormais fameuse DETR est devenue une manne précieuse, indispensable à la réalisation de bien des investissements municipaux, surtout lorsque certains conseils départementaux ne peuvent dégager un budget important d'aide aux communes. Or cette source de financement gagnerait à devenir un peu plus transparente. Certains orateurs ont évoqué feu la réserve parlementaire, stigmatisée, diabolisée, guillotinée pour crime de clientélisme. Celle-ci rendait pourtant bien des services, notamment aux communes peu fortunées et aux associations locales, dont nous connaissons tous l'importance pour entretenir le lien social. Nombreux sont aujourd'hui les parlementaires qui regrettent de l'avoir sacrifiée sur l'autel de la démagogie. Mais qu'est donc la DETR si ce n'est une gigantesque réserve préfectorale ? Cette distribution de subventions à la discrétion du préfet ne constitue-t-elle pas une forme de clientélisme ? Quand on met en parallèle les 130 000 euros annuels dont bénéficiaient nos collègues et les 15 millions d'euros que répartit le préfet de l'Oise, on voit toute la relativité entre le clientélisme parlementaire et l'influence préfectorale, dont personne ne peut nier le rôle politique. Qui mieux qu'un élu enraciné depuis des décennies connaît son territoire et ses habitants,

et de cohérence. Un préfet éclairé par la lanterne de celles et ceux qui ont, à la fois, la légitimité démocratique et la lucidité offerte par un fil d'Ariane local est toujours plus efficace, préférable et plus équitable.

des refus de DGE. La transparence est plus que jamais nécessaire, compte tenu des difficultés budgétaires des collectivités locales et des demandes légitimes des citoyens en matière de distribution et de redistribution de l'argent public. Quel

L'attribution de la DETR dépend uniquement du préfet du département. L'avis des parlementaires qui siègent dans les commissions DETR

est alors présenté à la commission DETR du département, dont l'avis est non pas consultatif, mais décisionnel. L'enveloppe de subventions au titre de la DETR que peuvent proposer les parlementaires du département ne peut pas être supérieure à 20 % de l'enveloppe totale. totale. Cela correspond peu ou prou au du montant de l'ancienne dotation parlementaire de 2017 et du montant de la DETR en 2020, soit, respectivement, 86 millions d'euros et un milliard d'euros.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.